mesdames, messieurs les députés et sénateurs, mesdames, messieurs les représentants du corps diplomatique, le moment est solennel, les circonstances inédites. Pour la première fois de notre histoire parlementaire, nous accueillons le président d'un pays en guerre, d'un pays dont la capitale est assiégée, sur lequel les frappes redoublent d'intensité en ce moment même. Car l'inadmissible est en train de se produire : la guerre en Europe, aux portes de l'Union européenne ; la guerre en Ukraine. Votre peuple, monsieur le président de l'Ukraine, force l'admiration. Alors qu'il est la cible d'une agression que rien ne peut justifier, alors qu'il est la victime d'un appétit de conquête territoriale qui fait voler en éclat toutes les règles de la communauté internationale, alors qu'il est la proie de la folie meurtrière des autorités russes, le peuple ukrainien se bat. Les Ukrainiens, civils et militaires, résistent jusqu'à l'héroïsme pour défendre la souveraineté de leur pays et leur liberté aux yeux de l'Europe et du monde. Je souhaite, mes chers collègues parlementaires, ainsi que les membres du Conseil de Paris, que je salue et qui nous écoutent, que nous nous levions et que nous applaudissions, afin de rendre hommage au courage du peuple ukrainien et au vôtre, monsieur le président.

Vous nous direz dans un instant, monsieur le président de l'Ukraine, ce que vous attendez de notre pays, la France. Permettez-moi de vous remercier d'avoir fait le choix, en pleine tourmente, de vous adresser aux parlements des grandes démocraties, singulièrement au Parlement français, pour transmettre le témoignage de l'Ukraine et vos attentes. Ne doutez pas de notre soutien, pour aujourd'hui et pour l'avenir

Monsieur le président de l'Ukraine, monsieur le président du Sénat, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les représentants du corps diplomatique, président de l'Ukraine, de vous accueillir au sein de l'Assemblée nationale. Nous connaissons votre attachement à la France, où vous avez effectué votre premier déplacement officiel à l'étranger après votre élection en tant que président de l'Ukraine. Vous aviez ainsi engagé, dès 2019, un dialogue fructueux avec la France. Je tiens également à saluer la présence parmi nous de l'ambassadeur d'Ukraine en France, M. Vadym Omelchenko. Depuis

Depuis maintenant près d'un mois de guerre, les Ukrainiens se battent et résistent de façon héroïque à l'agression militaire russe. Soyez sûr, monsieur le président, de la solidarité et de l'entière mobilisation de la représentation nationale. Nous continuerons de veiller à ce que tout soit mis en oeuvre pour vous porter assistance, qu'il s'agisse de l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'agresseur ou de la fourniture d'un soutien humanitaire aux Ukrainiens comme aux réfugiés. Nous avons tous vu ces images choquantes, bouleversantes, de villes ukrainiennes bombardées et assiégées. La France condamne ces actes et ces bombardements indiscriminés visant les populations civiles. Cela doit s'arrêter immédiatement et nous appelons la Russie à se conformer au droit international humanitaire. Dans ces circonstances tragiques, le peuple ukrainien fait preuve d'une résistance admirable. Je tiens à saluer son courage et celui des autorités ukrainiennes. Sachez que nous demeurons à vos côtés. Monsieur le président de l'Ukraine, vous avez la parole.

suis reconnaissant d'avoir l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui. Je suis sûr que vous savez très bien ce qui se passe en Ukraine, vous savez pourquoi cela se produit et vous savez qui est coupable, même ceux qui se cachent la tête dans le sable et essaient de trouver de l'argent en Russie. Je m'adresse à vous, qui êtes des gens honnêtes, rationnels et courageux,

Elle est morte. En Ukraine, en Europe, en 2022, pour des centaines de millions de personnes, il n'était pas imaginable que le monde puisse être détruit. Je vous demande d'observer une minute de silence en l'honneur et à la mémoire des milliers d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens qui ont été tués à la suite de l'invasion russe du territoire ukrainien.

Après des semaines d'invasion, Marioupol et d'autres villes ukrainiennes frappées par l'occupant russe rappellent les ruines de Verdun, voit sur les photos de la Première Guerre mondiale que chacune et chacun connaît. L'armée russe ne distingue pas les lieux qu'elle cible : elle détruit tout, les quartiers résidentiels, les hôpitaux, les écoles, les universités- tout. Elle brûle tout : les entrepôts de nourriture et de médicaments- tout.

que les soldats russes tuent sur les routes, des journalistes qu'ils tuent sachant exactement qu'ils sont des journalistes,

Tout cela a été bombardé par les troupes russes, écrasé par l'artillerie russe et brûlé par les tirs de missiles russes.

Vous savez ce que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Ces mots sont importants pour vous : je le sens et les Ukrainiens le ressentent. Nous attendons de la France, de votre leadership, que vous fassiez en sorte que la Russie cherche la paix pour mettre fin à cette guerre contre la liberté, contre l'égalité, contre la fraternité, contre tout ce qui a permis à l'Europe d'être Nous attendons de la France, de votre leadership, la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. On peut le faire ensemble.

Pendant la présidence française de l'Union européenne, une décision mûrie sera prise sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne : ce sera une décision historique à un moment historique, comme cela a toujours été le cas dans l'histoire du peuple français. Mesdames, messieurs les parlementaires, peuple français, demain, cela fera un mois que les Ukrainiens se battent pour leur vie et leur liberté et que notre armée s'oppose de manière héroïque

Pour que la liberté ne perde pas, elle doit être bien armée : chars, armes antichars, avions de combat, défense antiaérienne. Vous pouvez nous aider, nous en avons besoin. Pour que Pour que la liberté ne perde pas, le monde doit la soutenir avec des sanctions contre l'agresseur : chaque semaine, il faut un nouveau paquet de sanctions. Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe Renault, Auchan, Leroy Merlin et d'autres doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie, ils doivent arrêter de financer le meurtre d'enfants et de femmes, les viols

à l'avenir et à la façon dont nous allons vivre après la guerre. Il faut des garanties sûres, la garantie que la sécurité sera inébranlable et que la guerre ne sera plus possible dans ce monde.

comme la France a dit adieu au grand Belmondo. Merci à la France et gloire à l'Ukraine